Pendant des années, vous avez érigé le Sénat en contre pouvoir. Il nous faut avoir pleinement conscience de la situation. Depuis plusieurs mois, l’intervention du président Emmanuel Macron met en cause l’équilibre institutionnel de la République. Le Sénat est aujourd’hui utilisé pour dévoyer le bicamérisme et affaiblir le pluralisme. Les chiffrages fantaisistes pour décrédibiliser la censure, pourtant seule réponse possible au 49.3, et le contournement des discussions par l’adoption du projet de loi de finances (PLF) en commission mixte paritaire sont autant de coups de force. De fait, vous acceptez de contourner les débats à l’Assemblée nationale et, du même coup, la volonté des Français exprimée dans les urnes. C’est du jamais vu : l’Assemblée nationale n’aura à aucun moment discuté la seconde partie du budget Cerise sur le gâteau, le 1décembre dernier, une seconde délibération du Gouvernement balaie en quelques secondes des jours de travail sénatorial. Sont ainsi supprimés vingt sept amendements de justice sociale et fiscale adoptés par notre assemblée.

En effet, la reprise des débats sans interruption de la session parlementaire est contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 47 de la Constitution. Le Gouvernement devait présenter un nouveau projet de budget

Le peuple va t il se satisfaire longtemps de donner les pleins pouvoirs à un seul individu, et ce dans une confusion idéologique croissante et au cœur d’une crise sociale et démocratique ? Le peuple va t il se satisfaire de laisser les pleins pouvoirs aux milieux financiers et des affaires ? Attention, mes chers collègues, l’intérêt général n’est plus le produit d’équilibre garanti par le politique ! Un mur se dresse entre les populations et les lieux de décisions. C’est dans ces conditions que nous sommes parvenus au terme de l’examen d’un budget frappé d’un triple sceau

Les dossiers de surendettement des ménages explosent. Quelque 250 000 emplois industriels sont menacés dans notre pays. La productivité décroche et 15 % des Français sont en situation de grande pauvreté. Comment pouvons nous continuer à faire comme si de rien n’était ?

Où frappez vous ? Toujours là où le coup fait le plus mal ! Sur la santé, déjà exsangue, vous ôtez 250 millions d’euros. Nos hôpitaux suffoquent, nos soignants s’épuisent et vous leur demandez de se serrer encore la ceinture.

Parallèlement, les collectivités territoriales, qui forment pourtant le dernier rempart contre les fractures sociales et territoriales, subissent, encore et toujours, une nouvelle coupe. Derrière les grands discours, la droite sénatoriale n’a pas bronché. Allez donc l’expliquer aux citoyens et aux élus locaux ! Derrière chaque euro arraché aux collectivités, c’est la vie des gens qui est malmenée : factures qui explosent, salaires qui stagnent, services publics qui se délitent. Quand tout sera privatisé, nous serons privés de tout.

si vous êtes si prompts à couper dans les services publics, c’est pour mieux préserver un ordre de priorité, en érigeant en première place l’intérêt des grandes fortunes et des détenteurs de capitaux. Chaque année, 200 milliards d’euros sont versés aux entreprises sous forme d’aides publiques

de solidarité sur la fortune (ISF), symbole d’une fiscalité juste, plébiscité par 72 % des Français, qu’en faites vous ? La véritable cohérence de ce budget, c’est le rejet idéologique du partage des richesses. avez refusé de présenter un nouveau budget que les quelques timides mesures de justice fiscale du budget Barnier n’ont pas été reconduites. C’est pourquoi nous travaillons à utiliser tous les recours démocratiques et tous les interstices qui existent. Ce que nous voulons, ce sont des mesures pour que les Français vivent mieux. À la veille du probable coup de force de la commission mixte paritaire (CMP) sur le budget, nous déposerons, députés et sénateurs communistes républicains citoyens et d’outre mer un projet de loi d’urgence économique et sociale, sociale, pour répondre au chaos que vivent les Français au quotidien. Ce texte a été élaboré à partir des propositions des communes, des syndicats et des associations. Oui, la démocratie a encore une vitalité, une espérance un gouvernement devrait savoir la trouver. Cet élan démocratique se manifeste dans les communes, dans le mouvement social dans sa diversité, dans les entreprises, dans les territoires. mesures, dont l’abrogation de la réforme des retraites, le blocage des prix et de nouvelles recettes pour répondre à l’urgence sociale. Engagés au cœur de ce combat pour la démocratie et la justice, nous voterons résolument contre ce budget. Comme le dit André Chassaigne, qui aurait fait un très bon président de l’Assemblée nationale, « il faut révolutionner le lien entre la population et le pouvoir politique ».

de dépouillement de nos comptes publics et d’une flambée jamais atteinte de notre dette. Oui, la situation budgétaire de la France est catastrophique. Mais cette catastrophe n’a rien de naturel. Elle est le résultat d’un certain nombre de vos choix, d’une politique qui a favorisé les baisses d’impôts et les cadeaux fiscaux pour les plus fortunés, sans que les retombées économiques promises se concrétisent. Ces orientations ont été financées à crédit et nos comptes ont plongé dans le rouge. Au chaos de nos comptes publics s’est ajouté le chaos politique. Le texte sur lequel nous allons nous exprimer aujourd’hui a tout d’une création de Frankenstein. Ce budget, sur lequel pas moins de trois ministres de l’économie successifs se sont penchés, échappe à ses créateurs et plus personne ne sait qui en porte la réelle responsabilité politique, chacun tentant de faire oublier les causes réelles de la situation. Lorsque nous avons commencé nos débats à l’automne, le Gouvernement nous expliquait qu’il n’avait eu que quinze jours pour produire sa copie. Le Président de la République, plongé dans une forme de dilettantisme olympique, a fait le choix de prendre son temps – soixante jours exactement – pour nommer un Premier ministre. Ce budget a donc été réalisé à la hâte par Michel Barnier, qui s’est appuyé sur des prévisions de croissance et de recettes fiscales irréalistes, actant d’ores et déjà un recul massif pour l’État et les collectivités dans la conduite de leurs politiques publiques. Lors de nos discussions au Sénat, nous avions fait progresser la copie. Sans atteindre le niveau de justice fiscale dont notre pays a besoin, le débat sénatorial avait cependant produit du consensus sur un certain nombre de nouvelles recettes. Pourtant, à trois jours de sa censure, le gouvernement Barnier a imposé à la majorité sénatoriale,

exclusive du Rassemblement national pour ses négociations budgétaires. C’est ce choix irresponsable qui a abouti à sa censure. Malgré cette censure et ce revers démocratique flagrant, le troisième de l’année pour la ligne politique présidentielle,

Force a été de constater que la trajectoire budgétaire a primé sur notre trajectoire climatique. Devant le blocage et le dogmatisme de Bercy, confinant parfois au déni climatique et après une déclaration de politique générale qui a fait l’impasse sur le défi du siècle, les députés écologistes n’ont eu d’autre choix que de voter une première censure. Sénat. Privé de justice fiscale et de nouvelles recettes, le Gouvernement a choisi de brutaliser un peu plus le débat parlementaire. Des amendements de dernière minute ont fleuri sur beaucoup de missions budgétaires, déposés dans la nuit ou dans la matinée avant la séance, rabotant de plusieurs centaines de millions

Nous l’avons beaucoup utilisé ces derniers jours dans l’hémicycle, mes chers collègues, mais le terme de « rabot » est en fait impropre. Les coupes budgétaires n’ont pas touché tous les budgets de manière lisse et homogène. Des choix ont été faits. Certains budgets ont été préservés, d’autres, amputés gravement. Derrière l’apparence du rabot, vous avez en fait passé certains budgets à la tronçonneuse ! Des lois de programmation ont été préservées, pour la défense, la justice et l’intérieur. D’autres ont été sacrifiées, comme l’aide au développement ou la recherche. La copie finale que nous étudions est donc révélatrice d’un choix, celui de sacrifier l’avenir. À la lecture de ce budget tel qu’il ressort des travaux du Sénat, force est de constater que le déni climatique n’est pas l’apanage du président des États Unis. Il frappe désormais les deux rives de l’Atlantique. En dépouillant le budget de la diplomatie climatique, avec 35 % de crédits en moins pour l’aide publique au développement, en ruinant nos capacités de recherche, avec 630

par la petite porte budgétaire, vous êtes en train de faire sortir la France de l’accord de Paris, dix ans après l’avoir défendu. Pourtant, le dérèglement climatique frappe fort. Entre deux gouvernements, cet hiver, un département français, Mayotte, a été rasé par un cyclone, qui, comme d’autres catastrophes naturelles récentes, a mis en lumière à la fois les impacts climatiques dévastateurs de nos émissions et la vulnérabilité de nos territoires. La Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2024, a décrit de manière méthodique l’extrême vulnérabilité de notre pays aux aléas climatiques, qui vont se multiplier. les besoins d’investissement sont bien réels, vous faites le choix du déni. Même le budget alloué à la sécurité civile diminue de plus de 50 millions d’euros. Nous sommes aujourd’hui témoins de l’absence totale de vision stratégique face aux défis de notre époque. En désarmant fiscalement l’État, vous nous exposez au pire. La transition écologique n’est pas un luxe dont nous pourrions nous passer quelques années avant d’y revenir. Elle nécessite des engagements pérennes dans le pour que chacun y voie un destin commun. Quand les zones à faibles émissions, outils nécessaires pour la qualité de l’air, montent en puissance, vous décidez de sabrer massivement dans les aides au changement de véhicules, dans le soutien aux investissements pour les transports collectifs et dans le plan Vélo. La cohésion des territoires est fragilisée, vous aggravez les fractures sociales et territoriales tout cela va mal finir. Monsieur le ministre de l’économie, vous assumiez ce matin, dans, de rester droit dans vos bottes. En réalité, vous restez droit dans les bottes présidentielles, celles qui nous ont conduits dans l’impasse budgétaire, celles qui nous font courir dans le mur climatique, celles qui défendent une politique désavouée à de multiples reprises dans les urnes. Nous refusons cette marche forcée vers l’abîme. Nous voterons contre ce budget ! La parole est à M. Thierry Cozic, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. et Républicain. Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voilà réunis pour terminer l’étude d’un texte dont les conditions d’examen, pour le moins tumultueuses, ne reflètent que trop bien la situation politique dans laquelle nous a placés le Président de la République. Cet examen a été tumultueux, dis je, car, entre temps, le gouvernement qui défendait le présent budget a été censuré.

Un tel coup de force démocratique ne pouvait pas rester sans réponse. C’est tout affairé à négocier avec l’extrême droite que le Premier ministre Barnier s’est retrouvé trahi par sa partenaire de négociations qui n’en avait jamais assez. Un nouveau gouvernement est donc en place. Après avoir écouté la déclaration de politique générale qui, disons le franchement, s’apparentait plus à une déclaration d’inertie générale, je ne suis toujours pas rassuré. Je tiens à revenir sur le choix qui a été fait de reprendre la navette sur le budget d’un gouvernement que la représentation nationale a censuré. Ce choix, tout sauf anodin, n’est pas seulement dicté par des considérations de célérité budgétaire. Ce choix, d’apparence formelle, est profondément politique

bien plus véhément, profond, et qui à ce jour reste ignoré : le besoin d’alternance. C’est cette même demande d’alternance qui s’est fait jour lors des dernières élections législatives, que le Président a convoquées de son propre chef. Je le dis avec gravité : un changement de cap doit désormais s’opérer et être perceptible par tous. Avec Mélenchon ? Ce changement doit être radical, car la défiance envers le Président est énorme.

Je le redis, ne pensez pas que vous obtiendrez automatiquement notre clémence sur l’autel de la sacro sainte stabilité. La stabilité ne sera acquise qu’à la lumière de la légitimité des décisions que vous prendrez. C’est un fait : les sept années de politiques iniques et verticales du pouvoir macroniste ont été durement sanctionnées dans les urnes. Ce n’est pas parce que le Président utilise son pouvoir de nomination comme un pouvoir de décision que nous ferons comme si rien n’avait changé. Une fois de plus, la légitimité politique du Gouvernement qui se présente à nous est assise sur les trois formations politiques ayant perdu les dernières élections. Une telle analyse vous impose le compromis. Nous l’avons dit lorsque nous nous sommes vus, monsieur le ministre de

Ce constat s’impose à nous alors que, depuis la prise de fonction du président Macron, la rémunération des actionnaires a augmenté de 114 %, tandis que celle des dividendes a progressé de 46 % et celle des rachats d’actions de 286 %. Ces hausses astronomiques nous donnent le tournis.

le Trésor pour feuille de vigne. Bravo ! C’est pourquoi nous refusons ce budget d’austérité. Il n’est pas empreint de justice fiscale et il cherche, dans les poches de ceux qui n’ont pas créé le problème, une solution qui ne fonctionne pas.

En matière de justice sociale, le compte n’y est toujours pas non plus. Nous ne ferons pas les frais de votre incapacité à contenir vos partenaires Les Républicains, qui, hier soir, n’ont rien trouvé de mieux que de ne pas respecter l’engagement de leur Premier ministre sur la suppression de postes d’enseignants. Sur les retraites, je salue le retour au dialogue. Même si la mission flash que vous avez confiée à la Cour des comptes vous a permis de vous détourner ostensiblement du Conseil d’orientation des retraites (COR), je nous félicite du retour des partenaires sociaux sur l’injuste réforme des retraites de 2023. Un tel retour n’aurait pas été possible sans l’œuvre des socialistes et nous serons très exigeants sur les suites qui seront données à ce conclave. Nous resterons extrêmement vigilants, car nous avons pris l’engagement devant nos électeurs de ramener le scalp de la réforme des retraites.

Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, le compte n’y est pas. C’est pourquoi, dans les jours qui viennent, nous serons aussi vigilants qu’exigeants. Or les annonces perlées par voie de presse en forme de renoncements ne nous rassurent pas. rassurent pas. La dette est désormais un problème, mais le diagnostic est systématiquement mal posé, et ce sciemment puisque ce sont les services publics et l’État social qui se retrouvent sur le banc des accusés du déficit public. Ce budget ne fait qu’instruire une fois de plus un tel procès.

Lors des arbitrages que vous aurez à rendre prochainement, il vous faudra en tenir compte, sans quoi, je le dis très solennellement, au nom du groupe socialiste, et avec gravité : les mêmes causes produiront les mêmes effets.

le projet de loi de finances que nous devons voter aujourd’hui est sans doute le plus complexe de l’histoire de la V République. Ni les conditions budgétaires, ni les conditions politiques, ni encore moins les conditions médiatiques ne permettent un débat serein ou cohérent.

pour vérifier toutes ces informations ? Politiquement, ensuite, le pacte contre l’opinion conclu par certains partis et la personnalité d’Emmanuel Macron sont les seuls et uniques responsables d’une instabilité parlementaire, que nous n’espérons pas structurelle. Si ces partis sont parvenus à s’entendre pour sauver quelques prébendes, ils n’ont pu s’accorder pour construire un projet politique,

Ainsi, alors que les manques sont permanents et que les administrations comme l’économie se délitent, nous devons voter un budget pour économiser davantage. Nous avons proposé des économies. Elles reposent sur un principe clair : ne pas davantage écraser fiscalement la France qui travaille et celle qui souffre. Des agences trop nombreuses aux gabegies de notre politique migratoire, en passant par l’absence de contrôle d’opportunité ou de gestion, il n’y a malheureusement quasiment aucune rupture. Comme d’habitude, plus que l’arithmétique sénatoriale, c’est encore et toujours le conformisme et les œillères idéologiques qui ont bloqué ces mesures de bon sens. Néanmoins, si nos amendements n’ont pas été adoptés, certaines idées ont au Nous nous félicitons évidemment de la baisse des crédits pour l’aide publique au développement. Faut il rappeler que, en ces temps budgétaires difficiles, nous devons en premier lieu privilégier nos concitoyens et nos besoins, et non des financements dispendieux qui n’ont soutenu ni notre rang à l’étranger, en déshérence depuis sept trop longues années, voire davantage, ni notre économie ou nos partenariats Le choix du Gouvernement de recourir à des coupes budgétaires aveugles révèle deux choses : d’une part, des économies sont évidemment possibles ; d’autre part, ce gouvernement, comme les autres, refuse de faire de véritables choix politiques. En revanche, la décision du Sénat de maintenir la trajectoire de la loi de programmation militaire (LPM) est un signal positif, qu’il faudra défendre en commission mixte paritaire. Bien que nous considérions que certaines lois de programmation précédentes restent insuffisantes, un gouvernement responsable doit s’y tenir. En trois minutes, il me sera impossible de lister les manques du budget Barnier. Reste que de meilleurs choix étaient possibles, dans un temps aussi contraint que le vôtre et avec des équipes bien moins étoffées. Le contre budget du Rassemblement national, présenté par mon excellent collègue Jean Philippe Tanguy, répondait davantage à la double nécessité de baisser les dépenses publiques et de rendre aux Français leur argent, le tout avec une efficacité renforcée de nos services publics. Nous refusons en effet l’argument selon lequel on doit faire moins avec moins ou plus avec plus. Nous continuons de croire que nous pouvons faire plus avec moins, pour peu que l’on reconsidère les priorités. Il faut conclure. Il ne nous semble pas que tel soit le cas. Il y a une solution à la surenchère fiscale et à la purge sociale. En l’état, nous ne pouvons voter ce budget. La parole La parole est à Mme Vanina Paoli Gagin, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, le 10 octobre dernier, Michel Barnier déposait à l’Assemblée nationale un budget qu’il qualifia lui même d’imparfait, en laissant le soin aux parlementaires des deux chambres de l’améliorer.

Le débat désolant et la valse des milliards de taxes et d’impôts nouveaux adoptés laissaient le champ libre à notre chambre pour montrer son sérieux. du groupe Les Indépendants, nous avions estimé que ce projet de budget, certes perfectible, était un texte d’urgence pour éviter à notre pays une crise budgétaire d’ampleur. Malgré notre réticence naturelle à voter toujours plus d’impôts, nous avions accepté l’équilibre proposé par le Gouvernement, consistant à faire peser l’effort budgétaire, pour deux tiers, pour un tiers, sur une augmentation provisoire ciblée et très encadrée de la fiscalité sur les ménages les plus aisés et sur les plus grandes de nos entreprises. Ce budget devait également être l’un des premiers depuis quelques années à faire l’objet d’économies substantielles proposées par le Gouvernement. du groupe Les Indépendants, nous estimons que la baisse de la dépense publique est une absolue nécessité. Cette baisse, que nous promouvons, ne doit être ni brutale ni généralisée à toutes les compétences de l’État. En effet, celui ci doit impérativement continuer de financer ses missions régaliennes. Ces missions sont celles là mêmes qui justifient l’existence de l’État : assurer notre sécurité du quotidien ; rendre une justice impartiale ; nous protéger au delà de nos frontières avec une armée moderne, tout en assurant notre place dans le monde grâce à une diplomatie de premier rang. Voilà, mes chers collègues, quelle est la raison d’être de l’État. En plus de ses missions essentielles, l’État doit veiller à l’organisation de notre santé, de l’éducation de nos enfants, de la lutte contre le réchauffement climatique et, enfin, j’y reviendrai, il doit nous projeter dans l’avenir au travers de la recherche et de l’innovation, que nous souhaitons, nous aussi, sanctuariser. À cet égard, je me permets de déplorer que la loi de programmation pour la recherche n’ait pu être respectée dans ce projet de loi de finances. Mes chers collègues, je vous disais en introduction de mon propos que l’examen calamiteux du budget à l’Assemblée nationale avait laissé le champ libre à notre chambre pour montrer son sérieux. Qu’en a t il vraiment été ?

–, augmenté les impôts de production indirectement, la création d’un nouveau versement mobilité, et raboté le crédit d’impôt recherche, outil essentiel pour notre compétitivité et notre avenir.

La dégradation de la fiscalité, votée en première partie à rebours de l’effort accompli depuis 2017, a conduit notre groupe à s’abstenir sur le vote de ce texte.

et, surtout, sanctuariser ses dépenses d’investissement. En sacrifiant les dépenses d’avenir pour maintenir ses dépenses du quotidien, l’État ne se comporte pas tout à fait en bon gestionnaire. La baisse de l’investissement dans la recherche et l’enseignement supérieur, la baisse des crédits de France 2030 ou de ceux qui sont consacrés à l’écologie sont autant de renoncements à préparer l’avenir de nos enfants, pour financer les dépenses de fonctionnement de nos ministères. Mes chers collègues, nous avons devant nous deux potentielles crises budgétaires. La première, la plus lointaine, est le fruit de cinquante années ininterrompues de budgets en déficit. Cette crise budgétaire, nous le savons tous,

Nous mettrions l’ensemble de la machine de l’État en difficulté et nous plongerions alors nos concitoyens dans l’inconnu. Le groupe Les Indépendants ne souhaite pas ajouter une crise budgétaire à la crise politique que nous traversons depuis la dissolution. Nous savons que le propre des compromis

Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, chacun le sait, ce budget est celui de trois gouvernements : les premières négociations de préparation ont débuté au printemps, époque à laquelle Gabriel Attal était Premier ministre ; ce projet de loi de finances (PLF) a été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre dernier, date à laquelle Michel Barnier était Premier ministre ; après le vote de la motion de censure, ce sont les ministres du gouvernement de François Bayrou qui ont défendu les crédits des missions restant encore en discussion. Le texte que nous nous apprêtons à voter n’est ni le texte de Gabriel Attal, ni celui de Michel Barnier, ni celui de François Bayrou ; c’est celui du Sénat ! Celui du Sénat, et plus précisément celui de la majorité sénatoriale, car c’est un budget responsable. L’état catastrophique de nos finances publiques à la fin de l’été 2024 a obligé Michel Barnier à présenter une copie prévoyant un effort de 50 milliards d’euros, répartis entre 20 milliards de hausses de fiscalité temporaires et ciblées, et 30 milliards de baisses de dépenses. Le groupe Les Républicains a accentué cet effort en votant près de 3 milliards d’euros d’économies supplémentaires, dont 1 milliard au titre des agences et des opérateurs de l’État. Les travaux de la commission d’enquête demandée par notre groupe permettront de poursuivre ces mesures de rationalisation dans les prochaines années. assez rare pour être souligné, entre le vote de la première partie du PLF, le 1 décembre, et la clôture de la seconde partie, la nuit dernière, nos efforts ont permis de réduire le déficit public anticipé pour 2025 à hauteur de 0,1 point de PIB.

Sans les grandes collectivités, pas d’investissement public, outil indispensable à la vitalité économique de nos territoires. Nous offrons aussi la possibilité aux exécutifs locaux de lever des recettes supplémentaires, au travers de la hausse des droits Par ailleurs, les enquêtes d’opinion montrent que nos concitoyens attendent beaucoup de la police et de la justice. Un sondage datant du début de 2025 mettait en avant que, pour 70 % des Français, la lutte contre la délinquance était prioritaire, ce qui représente

L’augmentation des accises sur l’électricité à un niveau supérieur à celui qui prévalait avant la crise de l’énergie était inacceptable. C’était une mesure antisociale et anti écologique. Parce qu’elles auraient des effets délétères sur la croissance, le Sénat a rejeté toutes les hausses de fiscalité peu ciblées ; je pense, par exemple, à la hausse du PFU. Je l’affirme avec conviction : les mesures concédées par François Bayrou au parti socialiste ne sont pas des marqueurs socialistes. La majorité d’entre elles avaient déjà été portées par notre groupe et votées avant l’envoi de la lettre du Premier ministre à Olivier Faure

En commission mixte paritaire, les représentants du groupe Les Républicains veilleront à ce que la copie du Sénat ne soit pas dénaturée. La presse s’est largement fait l’écho de la sagesse sénatoriale, qui a refusé une baisse trop forte du budget du sport. Après la parenthèse qu’ont représenté les jeux Olympiques cet été, six semaines au cours desquelles nous avons réussi à faire nation autour de nos athlètes, il nous incombe de soutenir l’énergie positive véhiculée par le sport, alors que nos athlètes défendront les couleurs de la France à Milan Cortina

CumCum », contournement à grande échelle de l’impôt sur les dividendes. Il est temps de ne plus procrastiner sur cette question : notre assemblée vote en ce sens depuis 2019 Le vote de cette après midi n’est que le début d’un long chemin vers le redressement de nos finances publiques et la croissance durable. Cette semaine, la Commission européenne a validé la nouvelle trajectoire de nos finances publiques. Malgré une prévision de déficit en 2025 qui est désormais de 5,3 % du PIB, contre 5 % auparavant, et une croissance plus faible, nos partenaires européens ont décidé de maintenir leur confiance dans la capacité de notre pays à redresser progressivement la barre. Mais les efforts non faits cette année seront reportés sur les prochains exercices budgétaires, pour atteindre 3 % du déficit en 2029. atteindre 3 % du déficit en 2029. L’attractivité des nouveaux produits émis par l’Agence France Trésor, cette semaine, confirme la confiance retrouvée dans la dette française. Toutefois, ces efforts pris dans l’urgence ne sauraient suffire.

préempte l’avenir et l’adaptation de notre économie et de notre société à une France à +4°C. Dans les prochains jours, les discussions autour du financement de la sécurité sociale vont reprendre. Après l’État et les collectivités locales, la sphère sociale va devoir prendre sa part dans le redressement de notre trajectoire budgétaire. Des discussions sont ouvertes sur l’avenir du financement de notre système de retraite. Le cadre ouvert par le Premier ministre, à savoir une réforme à budget constant, laisse peu de marges de manœuvre, sauf à revoir l’architecture d’ensemble et l’articulation entre répartition et capitalisation. La situation appelle à des réformes d’ampleur, que nous attendons vainement depuis 2017. Le système de santé, la relation entre l’État et les collectivités, la fiscalité, la planification industrielle et écologique sont autant de priorités auxquelles nous devons répondre l’immédiat. Vous l’aurez compris, madame, messieurs les ministres, notre soutien au gouvernement auquel vous appartenez est un soutien vigilant et responsable. Dit autrement, le budget que nous allons voter est le plus mauvais budget, à l’exception de tous les autres

Monsieur le président, madame, messieurs les ministres,

À cette occasion, je tiens à souligner la qualité du débat budgétaire au sein de notre chambre, bien loin du tumulte de l’Assemblée nationale, auquel nos concitoyens, nos entreprises et nos collectivités ont assisté, Tandis que les extrêmes ont aboyé, la caravane de la dette a accéléré. Ils portent la responsabilité de la censure d’un gouvernement, des économies qui n’ont pu être réalisées, de l’absence de soutiens indispensables aux agriculteurs et de l’impossibilité pour les collectivités de financer des dépenses cruciales pour nos territoires. Nous saluons la méthode du Gouvernement : pragmatisme, dialogue, écoute et concertation avec l’ensemble des forces politiques, sociales et économiques. Celui ci a réussi à trancher le nœud gordien en trouvant un compromis avec d’autres forces républicaines pour proposer un budget à la France. Ce budget, s’il ne constitue qu’une première étape du travail de redressement de nos finances publiques, permettra enfin à la France de se doter d’un cadre budgétaire clair. Il contient des mesures qui, nous l’espérons, permettront de restaurer la confiance ainsi que la capacité d’action et d’innovation de nos entreprises et de nos concitoyens, où qu’ils se trouvent. Je pense notamment aux territoires ultramarins, qui bénéficieront de mesures concrètes, telles que l’exonération de l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) depuis et vers les départements d’outre mer, ou la baisse de TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, qui constituera un nouveau jalon dans le travail de lutte contre la vie chère. Nous nous félicitons de ce que le dialogue avec le Gouvernement ait permis l’ouverture de près de 500 millions d’euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement, destinés notamment à soutenir la reconstruction des territoires calédonien et mahorais, auxquels nous exprimons de nouveau tout notre soutien. Je pense également à nos concitoyens. Je salue, à ce titre, l’engagement transpartisan de notre assemblée en faveur du pouvoir d’achat des Français, notamment sur la baisse de 14 % des prix de l’électricité. Nous avons également répondu à leur demande de justice fiscale, grâce à des avancées comme le dispositif anti évitement sur les bénéfices des grandes entreprises et le relèvement du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF), une mesure portée par notre groupe. Le groupe RDPI a également œuvré pour répondre à leurs attentes sociétales en favorisant la sécurisation de la voie publique, par l’augmentation de la présence de la police nationale, et en soutenant l’économie, au travers d’un meilleur financement de la transition écologique de l’industrie. Nous saluons les avancées que ce texte apporte au secteur agricole. Le groupe RDPI y aura pleinement contribué, notamment au travers de l’amendement du président Patriat visant à aligner le régime fiscal des transmissions des terres agricoles et viticoles sur le régime commun des transmissions d’entreprises et, donc, à faciliter la transmission intergénérationnelle des PME familiales. De même, le nouveau crédit d’impôt « haies », introduit grâce à l’adoption de l’amendement de mon collègue Bernard Buis, favorisera la gestion durable des haies, donc celle des terrains agricoles. Enfin, nous sommes satisfaits du compromis qui a été trouvé concernant les efforts d’économies demandés aux collectivités. Initialement fixés à 5 milliards d’euros, ces efforts paraissaient trop importants au vu de la situation financière des collectivités. Ils ont donc été limités à 2 milliards d’euros, afin de maintenir la capacité d’investissement des collectivités et de leur permettre de dégager des marges de manœuvre supplémentaires. Malgré les avancées prévues dans ce PLF, nous devons rester vigilants. Le soutien du Gouvernement aux politiques sportives demeure à ce jour insuffisant. Notre groupe continuera de défendre l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques en commission mixte paritaire. Par ailleurs, attachés à la démocratisation culturelle, nous nous opposons évidemment à toute volonté de suppression du pass Culture, outil essentiel à la réduction des inégalités, que nous entendons préserver. De même, la situation budgétaire est particulièrement préoccupante, avec une dette publique de 3 303 milliards d’euros, un déficit prévu à 5,4 % en 2025 et un taux d’intérêt à dix ans de 3,40 %. Il est impératif de poursuivre l’assainissement de nos finances publiques et de dégager de nouvelles marges de manœuvre budgétaires. En l’absence de réserves, nous ne pourrons faire face aux prochains « cygnes noirs En dépit des défis qui restent à relever, ce projet de loi de finances pour 2025 constitue un premier jalon vers le redressement de nos finances publiques et la mise en place d’un cadre budgétaire plus juste et efficace. Grâce aux efforts conjoints du Gouvernement et de notre assemblée, ce texte porte des mesures concrètes et équilibrées, répondant aux attentes de nos concitoyens, de nos entreprises et de nos territoires. C’est pourquoi le groupe RDPI votera en faveur de ce projet de loi de finances, avec la conviction qu’il constitue une étape déterminante pour préparer l’avenir de notre pays.

l’arbitre a sifflé la fin du match budgétaire au stade du Luxembourg et le score s’affichera dans quelques instants sur le panneau lumineux à ma gauche ! Il a été marqué par une suspension de la partie de sept semaines, après l’éviction du sélectionneur Michel Barnier

Pour la fin de la deuxième mi temps, le sélectionneur a changé sa tactique de jeu, abandonnant une défense de fer pour laisser un peu d’espace à l’équipe adverse. Mais l’arbitre, M. Bercy, est toujours en place. Rien n’est joué. Si tous les observateurs prévoient une victoire au stade du Luxembourg, il faut prendre en compte le résultat du match aller au stade de la rue de l’Université.

et encore moins le résultat. Reste à espérer que le trophée sera remis sans avoir recours aux tirs au but ! Plus sérieusement, sur le fond, la seconde délibération

À l’issue de cette discussion budgétaire, certaines avancées sont bienvenues, comme l’allégement de l’effort demandé aux collectivités territoriales, qui passe de 5 milliards à 2,2 milliards d’euros, l’annulation de la suppression de 4 000 postes dans l’éducation nationale ou encore les mesures fiscales et budgétaires en faveur des outre mer. Une certitude persiste : le Gouvernement a, une fois de plus, malmené le Parlement et abusé du rabot budgétaire répondant à une logique de gestionnaire de court terme et non à la nécessité de construire la France de demain. Finalement, que restera t il des 3 831 amendements déposés lors de ce marathon budgétaire ?

Lors de la discussion budgétaire, le groupe RDSE a défendu une position responsable, avec des amendements de justice sociale, fiscale et territoriale visant à contribuer à la maîtrise des dépenses publiques et à la préservation du pouvoir d’achat des Français,, par exemple, la suppression de l’augmentation de la fiscalité sur l’électricité,

D’autres encore tendaient à réduire les doublons, voire les triplons, de dépenses administratives, sans tomber dans la logique « bercynienne » du rabot, tout en rationalisant la jungle des 438 opérateurs de l’État, qui mobilisent – rappelons le – 80 milliards d’euros Seule une dizaine de nos amendements ont été adoptés ; c’est une maigre consolation. Dans la partie recettes, la seconde délibération a supprimé l’amendement sur le PFU et celui qui visait à instaurer les taxes sur les bouteilles en plastique, nous privant de ressources utiles et pleinement justifiées, sans oublier mon amendement tendant à fiscaliser les automates de paiement, rejeté année après année. Dans la partie dépenses, je ne peux que me réjouir de l’élargissement du prêt à taux zéro. Mais la situation du logement reste dramatique : le compte n’y est pas. Or le logement, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), les investissements des collectivités locales et le taux de croissance sont autant de marqueurs déterminants pour la santé de notre économie, traduisant son dynamisme et le rythme des rentrées fiscales. Je suis inquiet, car ils seront pénalisés par ce budget pour 2025. Si je ne peux pas reprocher au Gouvernement de chercher à réaliser l’équilibre des comptes, je conteste certains de ses arbitrages. Aujourd’hui, seule la nécessaire maîtrise des finances publiques permettra à la France de regarder son avenir dans les yeux. Mais comment réussir ce tour de force en l’absence d’un plan pluriannuel de redressement des finances publiques, sans remise en cause des paradigmes de la présentation des crédits et des dépenses dans le budget, et sans l’instauration d’un dialogue sincère avec les collectivités locales et les organismes paritaires ? Alors que l’ADN du groupe RDSE est de faire avancer les débats sans dogmatisme pour créer du consensus, force est de constater que notre voix n’a pas été entendue. Loin d’être satisfait, mais considérant qu’il est nécessaire que notre pays soit doté d’un budget, je m’abstiendrai, comme la plupart de mes collègues du RDSE.

Vous le savez tous, la situation de nos comptes publics est particulièrement préoccupante, ce qui se traduit par un recours à l’emprunt qui commence à devenir extrêmement important.

plutôt que ces recettes hasardeuses, le groupe Union Centriste aurait préféré des recettes plus sûres. Une hausse de deux points du taux normal de TVA

de la seconde partie du texte, nous avons déposé des amendements visant à réduire des crédits sur à peu près toutes les missions de l’État, considérant qu’il importe de réaliser un effort de modération des dépenses publiques.

Merci,

Vos bulletins de vote personnels sont à votre disposition dans une enveloppe placée dans le tiroir de votre pupitre. Si vous êtes titulaire d’une délégation de vote, vous y trouverez également une enveloppe contenant les bulletins de vote de votre délégant.

au sort la lettre par laquelle commencera l’appel nominal. Le

Le scrutin est clos. Mme et M. les secrétaires vont procéder au dépouillement

Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons donc au terme de la discussion du projet de loi de finances pour 2025, qui s’est déroulée, chacun le sait, dans des conditions

Afin d’assurer la continuité de la vie de la Nation, nous avons été conduits à adopter définitivement, le 18 décembre 2024, le projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances Dans ce contexte particulier, nous avons de nouveau battu des records de durée d’examen et de nombre d’amendements. Nous avons débattu pendant 164 heures,

Le nombre d’amendements déposés a presque doublé en cinq ans. Cette tendance me conduit, mes chers collègues, à renouveler les interrogations que je vous livrais l’an dernier sur le nombre d’amendements et la possibilité de préserver la qualité de nos débats dans un cadre constitutionnel aussi contraint que

les 75 rapporteurs pour avis des autres commissions, ainsi que les présidents de ces dernières et les chefs de file des groupes politiques, pour leur contribution à nos débats.

au regard de la gravité de la situation, j’ai « mal à mon pays » ; je voudrais avoir une France plus rayonnante, celle qui a ébloui le monde lors des jeux Olympiques, plutôt que de devoir redresser la situation

Mme la ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs,

prendre en compte le plus grand nombre de ces priorités, dans le cadre, naturellement, des contraintes et des axes que nous avions choisis.

visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique est parvenue à l’adoption d’un texte commun. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi

impossible juridiquement que le Parlement, c’est à dire chacune de ses deux chambres, adopte le texte que nous examinons aujourd’hui. La véritable reprise de la discussion du PLFSS aura donc lieu en février prochain, lorsque l’Assemblée nationale examinera, en nouvelle lecture,

Sans aucune mesure législative ou réglementaire d’amélioration du solde, le déficit en 2025 pourrait atteindre environ 30 milliards d’euros et les déficits annuels pourraient encore augmenter d’ici à 2028. Cela ne sera pas soutenable.

et d’instaurer une revalorisation différenciée des retraites permettant d’économiser 2,6 milliards d’euros. Tout cela, vous le savez, a disparu avec la censure. Il prévoyait également d’instaurer une contribution de solidarité pour le travail.

de le faire pour celui de l’État. Nous le devons non pas seulement à ceux qui aiment la matière budgétaire, mais surtout et avant tout aux acteurs de notre système de protection sociale,

nous sommes réunis pour un exercice étrange et largement formel : voter les conclusions d’une CMP considérées comme rejetées par les députés à la suite de l’adoption d’une motion de censure, le 4 décembre dernier.

assurés, actifs, retraités, employeurs, acteurs de la sécurité sociale, professionnels de santé et gestionnaires des caisses de la sécurité sociale, tous étaient mobilisés –, d’autre part, la préservation des emplois et de la qualité des services. À ce titre, je tiens à revenir

il y a presque deux mois, le 26 novembre dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’est réunie. J’ai eu l’honneur d’y représenter notre groupe.

Malheureusement, l’irresponsabilité des députés de gauche et d’extrême droite en a décidé autrement. En votant en faveur de la motion de censure déposée sur ce projet de loi, les intéressés ont fait le choix d’aggraver la crise institutionnelle, économique et sociale que nous traversons. Si cette fin d’année a constitué une trêve bienvenue et si la loi spéciale du 20 décembre dernier garantit le versement des prestations, la sombre réalité de nos comptes sociaux n’a pas disparu par magie. Le déficit de 18 milliards d’euros des comptes de la sécurité sociale pour l’année 2024 nous le rappelle, tout comme les perspectives négatives pour les quatre années à venir. Il nous revient donc, plus que jamais, d’engager sans délai des efforts importants pour retrouver la maîtrise de nos comptes sociaux et pour ne pas laisser une dette insoutenable aux générations futures. du projet de loi au Sénat, le groupe RDPI s’était majoritairement abstenu, considérant qu’il subsistait quelques points de divergence importants, en particulier à l’article 6.

en compte. Le groupe RDPI soutient le compromis trouvé à l’article 6. Alors que le gouvernement Barnier souhaitait réaliser 4 milliards d’euros d’économies au travers de la refonte du système d’allégement des cotisations patronales, le texte de la CMP ramène l’effort à 1,6 milliard d’euros. Mes chers collègues, notre groupe a été le seul à défendre unanimement et à voter au Sénat la suppression de cet article. Au delà du risque de destruction de plusieurs dizaines de milliers de postes, revenir sur les politiques de soutien à l’emploi que nous menons avec réussite depuis 2017 était inconcevable, au risque d’effacer les succès obtenus sur le front du chômage. Au contraire, favoriser le travail et la compétitivité de nos entreprises c’est améliorer l’état de nos comptes sociaux. Le compromis trouvé en CMP sur cet article est donc une bonne nouvelle pour l’emploi.

Si le texte de la CMP nous paraît très acceptable, les députés repartiront néanmoins la semaine prochaine de la version du Sénat. Par ailleurs, nous accueillons avec enthousiasme la récente annonce du Premier ministre de rehausser les dépenses de l’Ondam pour 2025 de 3,3 % par rapport à 2024, au lieu des 2,8 % envisagés, afin de soutenir l’hôpital, qui en a bien besoin. Je salue aussi l’annonce d’un Ondam pluriannuel – il était temps ! Comment, en effet, réformer notre système de santé sans vision politique, qui impose de regarder loin tout en agissant vite au service de nos concitoyens, de leurs médecins et de leurs soignants ? Mes chers collègues, ce PLFSS n’est ni un simple exercice comptable ni une guerre entre branches, les unes que les autres. Il s’agit avant tout d’un véritable contrat social, qui doit nous engager et incarner notre devoir de garantir l’équité médico sociale sur l’ensemble de nos territoires.

comme sur le PLFSS, notre groupe est ouvert à plus de justice sociale et à une meilleure protection de nos concitoyens, tout en prenant garde à la soutenabilité budgétaire. Je répète en cet instant, avec gravité, que les Français nous demandent de nous retrousser les manches et de travailler ensemble au service de l’intérêt général, sans sectarisme. Alors, plus que jamais, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, faisons enfin preuve de responsabilité. Pour notre part, nous y sommes prêts !

il y a deux mois, presque jour pour jour, j’entamais mon explication de vote sur le PLFSS en affirmant que l’inédit devenait la norme. Je ne croyais pas si bien dire ! Le lendemain, le 27 novembre, un accord en commission mixte paritaire était trouvé – une première depuis

Notre groupe partage le souhait du Gouvernement d’écourter cette période d’incertitude et d’instabilité en repartant non pas d’une feuille blanche, mais des débats précédemment menés au Parlement. Même si cet exercice nous contraint à discuter d’un texte déjà obsolète, il nous permet également,

la méningite dans les collèges. Les efforts de pédagogie doivent être renforcés, y compris sur la grippe, qui connaît un pic de mortalité effarant cette année – on pourrait atteindre les 10 000 morts ! Ce coût humain ainsi que les fortes tensions qu’il engendre à l’hôpital sont à mettre en regard du faible coût financier de la vaccination. Nous devons être plus convaincants sur ce dernier sujet, y compris chez les soignants, qui se protègent peu. L’obligation ne doit pas être un tabou ; à titre personnel, j’y suis favorable. Nous souhaitons également maintenir les mesures en faveur de la santé sexuelle, comme la généralisation des centres spécifiques, la meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap et l’expérimentation visant à rembourser, avant le dépôt de plainte, les tests et analyses de détection de soumission chimique. Nous travaillons sur ce dernier point au sein d’une mission gouvernementale. Nous soutenons certaines mesures qui permettent d’améliorer l’offre de soins, comme la lutte contre les rendez vous non honorés et l’exonération de cotisations d’assurance vieillesse pour les médecins libéraux en cumul emploi retraite. La généralisation de l’expérimentation permettant aux infirmiers de signer des certificats de décès est une excellente mesure, que nous appelons de nos vœux depuis plusieurs années. Enfin, je veux mentionner la question du financement. Travailler sur la pertinence des prescriptions est essentiel, mais

souscrire. Toutefois, ne nous y trompons pas : sans vision pluriannuelle, sans stabilité, sans réforme structurelle, le répit sera de courte durée.

de la sécurité sociale continue de reposer presque exclusivement sur les actifs, dans un contexte de baisse de la natalité et de hausse du coût de la santé, il nous faudra ouvrir sans tabou ni posture dogmatique le chantier du temps de travail et de l’employabilité des seniors,

tout le moins, si les Français travaillent plus, il faut les payer plus. Nous souhaiterions également aller plus loin sur la fiscalité comportementale, notamment sur les produits transformés tels que le tabac et l’alcool. J’insiste personnellement sur l’alcool, dont les conséquences demeurent un tabou dans le pays du vin, alors qu’il cause 41 000 décès et coûte 102 milliards d’euros par an. Voilà un moyen de mieux prévenir les maladies, de baisser nos dépenses et d’augmenter nos recettes poursuivre la navette parlementaire et d’aboutir à l’indispensable adoption du budget de la sécurité sociale pour 2025, notre groupe ne s’opposera pas à ce texte. Nos voix se répartiront entre abstention et vote en faveur du projet

longtemps. Pourtant, reconnaissons que nous n’avons pas pu nous réjouir très longtemps, car les germes de la censure apparaissaient à l’intérieur même de la commission. Je ne referai pas le match, d’autant que le PSG a gagné le sien hier… Au fond, le gouvernement Barnier est tombé pour avoir tenté de réguler nos dépenses sociales

finances. Faisons en sorte que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Le PLFSS est un texte essentiel, parce qu’il est l’un des piliers, peut être même le pilier

ou famille. En tant que rapporteur pour cette dernière, permettez moi de m’inquiéter de la nouvelle baisse de notre natalité : 663 000 bébés sont nés en France en 2024, soit 2,2 % de moins qu’en 2023 et 21,5 % de moins qu’en 2010. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit maintenant à 1,62. Ces chiffres doivent nous alarmer, mais, au fond, sont ils si surprenants ? J’ai bien conscience que les causes sont multiples, notamment l’anxiété qui règne et qui est propagée dans la société française. Affirmons le clairement : notre politique familiale n’est pas à la hauteur des enjeux. S’ajoutent à la fin de l’universalité des allocations familiales, décidée en 2015, la crise des modes de garde et la difficulté croissante pour les familles de trouver une place en crèche ou une assistante maternelle. En réalité, il est urgent de revisiter du sol au plafond notre politique familiale. Mes chers collègues, les défis posés par le PLFSS 2025 sont nombreux. Pour y répondre, Élisabeth Doineau et Philippe Mouiller ont déjà évoqué les pistes du Sénat – je n’y reviendrai pas. Nous n’aurons d’autre remède

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’exercice auquel nous nous livrons aujourd’hui est particulièrement affligeant, symptomatique de la situation politique que nous sommes en train de vivre. Plutôt que de respecter le vote des Françaises et des Français lors des élections législatives anticipées de juin dernier, où la gauche est arrivée en tête en nombre de députés, ne vous en déplaise, le Président de la République préfère nommer des Premiers ministres issus de sa minorité parlementaire.

À son arrivée, le gouvernement Bayrou, pas plus légitime que le précédent, avait deux options. La première consistait à écouter le peuple et ses représentants parlementaires en déposant un nouveau budget de la sécurité sociale, qui prenne en compte la situation de notre système de santé, qui abroge la réforme des retraites, qui mette à contribution les superprofits, etc. La deuxième option consistait à faire l’autruche en reprenant le projet de loi du gouvernement Barnier. C’est évidemment ce choix qui a été fait.

Dans la saison 1,, le gouvernement Barnier a joué le chrono en déposant un certain nombre d’amendements pour empêcher l’examen du texte

heures gratuites pour financer prétendument le grand âge, suppression de l’indépendance du service de contrôle médical de l’assurance maladie et enfin étalement de l’augmentation des cotisations sociales des hôpitaux et des collectivités sur quatre ans au lieu de trois. Je parle, évidemment, de la CNRACL. Dans la saison 2,, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord pour la première fois depuis quinze ans entre les deux chambres. Les députés et sénateurs se sont accordés sur les 130 articles restant en discussion en supprimant la journée de sept heures et en réduisant les économies

La ministre des comptes publics a confirmé que « travailler sept heures de plus par an, dès cette année, pour financer la dépendance des personnes âgées était une piste sur la table ».

il a beau être conscient qu’il devrait prêter attention aux mystères qui se déroulent là bas sur la scène, il n’arrive pas à rester éveillé. » Comment ne pas le comprendre, ce citoyen peint par Walter Lippmann

Le 4 décembre dernier, dans un coup de tonnerre pourtant bien prévisible, l’Assemblée nationale rejetait ce texte. Du même coup, elle faisait tomber le gouvernement de Michel Barnier, acoquiné dès ses commencements à l’extrême droite, lui confiant même son destin. Quelle leçon pour vous, monsieur le ministre ! Aucun démocrate ne peut accorder ne serait ce qu’une once de confiance à la parole de l’extrême droite. Si l’on fait l’erreur tragique de la croire, aussitôt elle n’hésite pas à baisser le pouce dans une forme d’exécution publique et à détruire brique par brique nos institutions. L’extrême droite ne dit jamais son nom véritable. Quand l’un de ses émissaires montre le bout de son nez, on dit : « C’est elle, vous croyez ? Il ne faut rien exagérer… » Puis un jour, cet émissaire accède au pouvoir et un salut nazi fait de nouveau la une des journaux. Ne l’oubliez pas : le projet du Gouvernement pour le budget de la sécurité sociale ne doit rien devoir à l’extrême droite. Les Françaises et les Français l’ont clairement exprimé lors des dernières élections législatives aucune compromission, aucune rupture du cordon sanitaire, aucune trahison du mandat populaire. Dès lors, vous n’avez d’autre choix que de vous tourner vers les forces républicaines, notamment vers la gauche et les écologistes.

D’abord, parce qu’il comporte des mesures antisociales que nous rejetons, au premier rang desquelles la désindexation – certes partielle – des pensions de retraite sur l’inflation,

; nous serons attentifs à ce qu’elles soient maintenues au cours de la navette parlementaire. Je pense à la réforme des exonérations de cotisations sociales, au dispositif Handigynéco, à l’annualisation du rendez vous « M’T dents », à la réforme de Mon soutien psy. En conclusion, le destin de ce texte rappelle que l’avenir du budget de la France, comme celui de la sécurité sociale, ne se fera que dans un esprit de parlementarisme éclairé par la démocratie sociale.

Le nouveau gouvernement Bayrou est alors nommé, issu une nouvelle fois d’une formation partisane minoritaire. M. Bayrou s’appuie, lui, sur le front républicain et invite à des négociations avec les groupes parlementaires socialiste, communiste et écologiste afin de faire adopter un budget pour pour l’État et la sécurité sociale. Les discussions s’engagent et doivent continuer. Les socialistes resteront ouverts, mais exigeants pour adopter des mesures qui changeront le quotidien des Français. Les échanges avec le groupe socialiste ont mené à la remise en question de la réforme des retraites de 2022, impopulaire auprès de 93 % des actifs. Le sujet est enfin sur la table des négociations du Gouvernement avec les partenaires sociaux. Nous leur faisons confiance pour trouver une issue favorable avant le retour d’un nouveau texte au Parlement.

prévus. Je tiens à alerter sur l’incapacité financière des hôpitaux à assumer les hausses de cotisations CNRACL. Nous avons noté l’abandon des déremboursements des consultations et des médicaments, mais nous ne sommes pas dupes : les mutuelles ont anticipé des augmentations de tarifs. À la fin, c’est toujours le malade et l’assuré qui

2025, ce qui nous a conduits à voter contre le budget. La répétition de ce scénario sur le budget de la sécurité sociale ne saurait nous satisfaire. Nous ne pouvons accepter des coupes budgétaires sur l’hôpital, sur l’autonomie des personnes âgées des personnes âgées ou handicapées, sur l’enfance… Le Gouvernement ne peut pas reprendre d’une main ce qu’il vient de donner de l’autre. Concernant les recettes, nous attendons des signes remarquables, qui démontreraient enfin votre attachement à la justice sociale et fiscale,

doit être une priorité. Il est de notre devoir de protéger les Français de ces dérives. Enfin, la préservation de notre système de sécurité sociale ne peut être efficace qu’avec des financements justes et pérennes. C’est pourquoi nous réaffirmons nos exigences pour une fiscalité plus juste. Le gouvernement Barnier avait ouvert la voie à une réduction des exonérations de cotisations inefficaces pour l’emploi et la compétitivité des entreprises. Nous ne renoncerons pas à aller chercher des recettes qui manquent cruellement à notre sécurité sociale. Pour préserver le budget de cette dernière, nous devons nous projeter dans une trajectoire de retour à terme à l’équilibre. La fuite en avant n’est pas une solution. Nous continuerons donc à proposer une fiscalité proportionnelle aux moyens de chacun. Nous nous opposerons fermement à la création d’une nouvelle journée de solidarité. La finance et le capital doivent contribuer à l’effort, au même titre que le travail. Monsieur le ministre, le sort de ce texte, issu de la commission mixte paritaire, importe peu. Je vous appelle donc à préparer avec nous un budget raisonnable

public de 3 200 milliards d’euros, avec une dette de 55 milliards en 2025. Pour la sécurité sociale, le déficit s’élevait à 16 milliards d’euros pour 2025, malgré les économies.

le coût de la fraude à la carte Vitale. Le maintien du déficit à 16 milliards d’euros de la sécurité sociale avec une désindexation des retraites, en préservant les petites pensions, n’a plus lieu d’être. Il nous faudra donc trouver

donner, notamment à nos agences régionales de santé et à nos établissements, une lisibilité sur plusieurs exercices budgétaires qui permette d’avoir une vision plus large et de définir des priorités. Il faudra naturellement protéger les piliers de notre système de santé, protéger les Français.

à nos élus locaux. Pour avoir été maire pendant plus de vingt ans et président d’une intercommunalité, je crois que les élus locaux doivent aussi pouvoir peser sur les décisions

conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 dans la rédaction résultant du texte